La séance est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance.- Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance. Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l'article 1 AA. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la prise en compte des inégalités territoriales dans la répartition des moyens du service public de l'éducation constitue une avancée importante. Le territoire de Wallis-et-Futuna souffre quotidiennement de son éloignement, de son isolement, de son enclavement, et les conséquences sont très handicapantes pour le fonctionnement de l'éducation : difficultés dans les déplacements, coût élevé des transports, aussi bien des personnes que des biens. Le coût des importations, et elles sont nombreuses, qu'il s'agisse de matériel pédagogique, de machines-outils, de matériaux de construction, est supérieur au minimum d'un tiers, et parfois

Il n'est pas étonnant de constater le manque de matériel, des outils dangereux ; par ailleurs, certains locaux ne répondent plus aux normes de sécurité, parce que dégradés ou vétustes. Les conséquences sont désastreuses pour ce qui concerne les résultats scolaires et l'atteinte des objectifs qui En 2017, les élèves en section CAP mécanique n'ont pas pu suivre de toute l'année la formation pratique que comporte l'enseignement de leur spécialité manque d'outils, retard des commandes et défaillances du point de vue de la sécurité des machines et des locaux ; c'est un enseignement au rabais. Monsieur le ministre, à Wallis-et-Futuna, l'enseignement est de la responsabilité financière de l'État.

En tant que président de la commission de l'aménagement du territoire, je regrette souvent que les politiques publiques ignorent la dimension territoriale. Cette initiative me paraît donc donc très opportune. Bien sûr, la finalité de l'école n'est pas l'aménagement du territoire. Mais nous savons tous que l'existence d'une école dans les territoires est un élément important

Robert. « Faire partager » les valeurs de la République ne se décrète pas. En outre, le partage de ces valeurs implique de les expliquer aux élèves, afin que ceux-ci en aient une compréhension réelle. Cette précision, qui revient à faire oeuvre de pédagogie, ce que font beaucoup d'enseignants à l'heure actuelle, permettra à la fois que ces valeurs soient mieux appropriées,

En outre, vous le savez, les programmes d'enseignement moral et civique prévoient déjà, dès l'école primaire, la présentation

2018, de 2019 et des suivantes, nous créons des postes à l'école primaire en France. Et cette création de postes nous permet non seulement de dédoubler des classes en REP et en REP+, mais aussi de défendre l'école primaire rurale. Il n'y a jamais eu aussi peu

peu de fois dans notre histoire. Cela nous renvoie au problème beaucoup plus important- j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans cet hémicycle -de la démographie en milieu rural, et plus généralement, de la démographie française,

à l'autre. La défense de l'école primaire rurale peut passer par différentes stratégies qui doivent être déterminées avec les maires, avec les élus locaux. Tel est le sens de la politique menée. C'est une politique du dialogue.

entre les élus locaux et l'éducation nationale, pour le rebond démographique et pour le rebond de l'école, et je suis à ce rendez-vous. Je tiens autant à l'école primaire rurale que chacune et chacun d'entre vous, et je ferai

M. le ministre a insisté sur un certain nombre de difficultés auxquelles notre école se heurte. Parmi elles figurent les inégalités sociales et, dans certains établissements,

disposition serait de nature à porter atteinte à la liberté d'organisation des établissements privés, laquelle procède de la liberté d'enseignement. En outre, des mécanismes incitatifs

pour des raisons qui ont été très bien rappelées. Cela étant, cet objectif figure déjà dans la loi : l'article L. 442-20 du code de l'éducation précise que l'article L. 111-1 du même code est applicable aux établissements d'enseignement privés qui sont associés au service public par contrat.

l'histoire de est complexe, multiple, polyphonique. Chant de guerre, elle fut aussi un chant révolutionnaire adopté par des peuples qui se réclamaient de « l'étendard sanglant » du premier couplet. Chacun et chacune se l'approprie selon sa culture personnelle, les circonstances particulières de sa vie ou sa tradition politique. Personnellement, je ne peux la chanter sans penser à celles et ceux qui l'érigèrent en arme de résistance, sur les Champs-Élysées, le 11 novembre 1940. novembre 1940. Dans les rangs de ces résistants de la toute première heure se trouvaient des gaullistes, des communistes, des socialistes, des chrétiens. Plusieurs d'entre eux connurent peu après la déportation et la mort. Ils incarnaient l'esprit de la Résistance et notre attachement collectif à la République, au-delà de nos origines et de nos sensibilités politiques ou philosophiques. Alors que est aujourd'hui le plus souvent entendue par les jeunes dans les enceintes sportives, je me demande comment il est possible de restituer, dans une classe, par une simple affiche, toute sa valeur symbolique et sa profondeur historique. Relisez les programmes : vous constaterez que et la devise républicaine sont régulièrement enseignées dans plusieurs matières et à plusieurs niveaux. Le corps enseignant n'a pas besoin d'une injonction, d'un affichage obligatoire, pour être pleinement investi dans sa mission d'éducation civique. Il faut lui faire confiance pour trouver les mots et les circonstances les plus appropriés, afin d'évoquer toutes les dimensions de notre hymne républicain.

pour le peuple », conformément à l'article 2 de la Constitution de 1958 : cette mention doit absolument figurer sur notre affiche ! Vous me permettrez de remarquer qu'aujourd'hui le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple est une forme de populisme qui devrait bien

notre credo. Parce qu'elles sont indispensables à la création et au renforcement du lien social, la liberté, l'égalité et la fraternité sont des valeurs que tous les élèves doivent assimiler dès le plus jeune âge.

Partant de ce principe, cet amendement vise à étendre l'obligation d'affichage du drapeau tricolore, du drapeau européen et des paroles du refrain de l'hymne national dans les salles de classe aux établissements des premier et second degrés privés hors contrat. En effet, le dispositif actuel ne s'applique qu'aux établissements publics et privés sous contrat. Or les valeurs et symboles de la République concernent l'ensemble des élèves et de la communauté éducative, quel que soit l'établissement scolaire fréquenté : la République doit s'imposer à tous

sur un sujet analogue, le législateur avait choisi, en 2013, de limiter l'affichage obligatoire des emblèmes et de la devise de la République sur la façade des établissements aux seuls établissements publics et privés sous

à partir du CE2 dans les programmes d'enseignement moral et civique. Dans une autre vie, j'ai un peu participé à leur écriture ; mes chers collègues, je vous propose de les lire

partager les valeurs de la République, y compris avec les élèves des écoles hors contrat. C'est pourquoi j'émets un avis favorable sur cet amendement n° 236. Cette disposition ne me paraît pas du tout contraire à la liberté de l'enseignement, puisque les textes prévoient déjà

et de. Les fondamentaux de la République ne sont pas négociables, quel que soit l'établissement, fut-il hors contrat, et la liberté d'enseignement ne doit pas s'arrêter aux portes de la République. Nous tenons donc fortement à ce que cet amendement soit adopté.

quelque chose de très réussi qui rassemblait la devise républicaine, l'hymne et le drapeau. Nous pourrons en tout état de cause proposer à chaque classe de France une affiche

Cet amendement vise à étendre l'obligation d'affichage du drapeau tricolore et du drapeau européen sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré aux établissements scolaires privés hors contrat, la disposition actuelle ne s'appliquant qu'aux établissements scolaires publics

faire une distinction entre les écoles publiques et les écoles privées hors contrat, lesquelles répondent à l'obligation d'instruction, mais ne participent pas au service public Je me suis déjà exprimé sur la liberté d'organisation de ces établissements. L'affichage sur leur façade des symboles de la République pourrait créer une confusion

Françoise Laborde, pour explication de vote.

et privés sous contrat, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Nous pensons utile que soit affichée de la même façon et dans les mêmes locaux et dans les mêmes locaux la charte de la laïcité à l'école. Il ne faut pas oublier que la France est une République laïque, et que la mission du service public de l'enseignement scolaire, à laquelle participent les écoles et établissements publics, mais aussi le secteur privé sous contrat, doit être guidée par le principe de laïcité. Pour les élèves, ce principe impliquant la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire et d'exprimer ses opinions dans les limites imposées par l'ordre public est souvent un concept un peu abstrait.

mise en place du Conseil des sages de la laïcité, avec des équipes nationales et académiques. Vous ne serez donc sans doute pas opposé à ce que la charte de la laïcité à l'école, antérieure à ces nouveaux organes, puisqu'elle date de 2013, soit apposée dans les locaux des établissements.

comme garant à la fois des libertés individuelles et des valeurs partagées d'une société qui dépasse et intègre ces différences pour construire un avenir

par l'explicitation qu'elle a permise de principes et par l'utilité qu'elle a depuis qu'elle est affichée dans les établissements publics. Comme il a été souligné, nous avons pris des mesures supplémentaires qui vont dans la même direction. Je suis toujours très attentif, chaque fois que je visite une école ou un établissement, à la présence de la charte de la laïcité. C'est une

madame la présidente.

permettez-moi de vous citer la lettre adressée aux instituteurs par Jules Ferry pour leur expliquer pourquoi la loi du 28 mars 1882 instituait l'enseignement moral et civique : « On n'a pas songé à vous décharger de l'enseignement moral : c'eût été vous enlever ce qui fait la dignité de votre profession. Au contraire, il a paru tout naturel que l'instituteur, en même temps qu'il apprend aux enfants à lire et à écrire, leur enseigne aussi ces règles élémentaires de la vie morale qui ne sont pas moins universellement acceptées que celles du langage et du calcul.

que cette affirmation est parfois discutée. Néanmoins, et même si ce sont des notions un peu absolues, auxquelles on n'accède jamais vraiment de manière totale, il est souhaitable que nous fassions tendre les enfants vers elles. Oui,

dont tous les autres découlent. L'école de la République doit évidemment dispenser un enseignement moral et civique ; la dimension morale appuie la dimension civique, comme la dimension civique soutient la dimension morale.

le respect de l'autre, ce n'est pas le bien ou le mal : c'est la déclinaison de la fraternité qui figure dans la devise républicaine. Le point d'appui est non pas le bien, mais les valeurs de la République qui se déclinent dans l'action de chacun.

en soi, qui ne puissent pas être interprétées selon les lieux et les périodes

quand des gamins ne sont pas suivis par leurs parents, ce ne sont pas les professeurs qui pourront leur inculquer la totalité des valeurs dont ils ont besoin pour s'insérer dans la société. Néanmoins, je suis convaincu que l'école doit transmettre non seulement le savoir,

ayons des racines judéo-chrétiennes semble atroce à certaines et certains d'entre vous, mais telles sont notre réalité et notre histoire ! Ensuite, des sédiments d'autres valeurs se sont ajoutés, mais notre école doit transmettre des valeurs, et la morale doit y avoir toute sa place

tendant à imposer l'installation dans les classes d'une carte représentant la métropole et les territoires d'outre-mer. Cette disposition, introduite dans l'article 1 B, a été supprimée par notre commission. Devant les

Les populations d'outre-mer, qui représentent entre 2,5 et 3 millions d'individus, sont purement et simplement ignorées, ce qui crée localement un sentiment de discrimination. À juste titre : apprendre

de permettre une représentation des territoires d'outre-mer, dès lors qu'une carte de France est affichée en salle de classe, sans pour autant exiger la présence systématique d'une carte de la France dans toutes les classes.

En tout cas, dans une salle de classe où l'on enseigne l'histoire et la géographie, il me paraît normal qu'il y ait systématiquement une carte

légiférer. La loi doit-elle définir tout ce qui doit être apposé sur les murs ? La manière dont on doit placer les cartes ? Doit-on dire aux professeurs d'histoire-géographie qu'ils doivent afficher les cartes de la France et les autres cartes ?

avec tout ce qui fait ses valeurs, avec l'ensemble de ses territoires ! C'est horrible ! Je ne comprends pas quand on sait, mon ami Karam l'a souligné, que 90 % de la biodiversité française

Souvent, les enseignants d'histoire ne savaient même pas comment avaient été construits les outre-mer ! Il a fallu une loi- du reste, nombreux ont été celles et ceux qui l'ont commémorée dans le jardin du Luxembourg, il y a quelques jours -pour graver dans le marbre que l'esclavage est un crime contre l'humanité.

Il faut en finir une fois pour toutes ; c'est une question de bon sens et c'est tout à l'honneur de la France, dans son immensité, dans sa dimension multimondiale.

Le jeune sénateur et vieux professeur d'histoire-géographie que je suis peut lui assurer que l'immense majorité des cartes de France

libellé : La parole est à Mme Marie-Pierre Monier. Les séances d'information et d'éducation à la sexualité dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées doivent permettre de faire reculer les violences sexistes et sexuelles, afin de véritablement contribuer à la lutte contre ces violences et de promouvoir effectivement une vision égalitaire entre les femmes et les hommes. L'âge moyen auquel se fait une première visite sur un site pornographique est de 14 ans et 5 mois, selon une étude de l'IFOP. Il s'agit là de visites volontaires, mais si nous parlons d'exposition à des images pornographiques, un enfant a en moyenne 11 ans lorsqu'il est exposé pour la première fois à du contenu pornographique en ligne, selon une enquête conduite par l'association Ennocence. Sont notamment en cause les fenêtres pop-up, les publicités ou le visionnage forcé par une tierce personne. L'exposition à ces images n'est pas sans conséquence, les enfants et les adolescents ayant du mal à prendre de la distance avec celles-ci. Comme le souligne le docteur Laurent Karila, psychologue et spécialiste de l'addiction sexuelle, cela génère des traumatismes. Visionner une scène pornographique à un âge très précoce- 7 ou 8 ans -est psychiquement similaire à un abus sexuel, à cause de la violence des images. Le visionnage de scènes pornographiques a aussi une incidence sur la construction de la sexualité. Selon le sondage de l'IFOP, près d'un adolescent sur deux a tenté de reproduire des scènes vues dans des films pornographiques. Au-delà des pratiques, les élèves visionnant ces images intériorisent les rapports de force et des stéréotypes dégradants pour les femmes. Les femmes sont très souvent représentées comme des objets et leur « non » signifie un « oui ». L'exposition précoce à la pornographie favorise donc la culture du viol. Les élèves concernés par ces séances sont de plus en plus exposés, et ce de plus en plus jeunes, à des images violentes qui peuvent les traumatiser et influencer leur comportement. Face à la diffusion de ces images, les établissements scolaires sont des lieux privilégiés pour déconstruire ces contenus violents et lutter contre la reproduction des violences sexistes et sexuelles. En informant et en sensibilisant les élèves, on peut aussi les avertir. Si jamais ils sont victimes ou témoins de tels comportements, ils sauront que ces actes sont à dénoncer et ne sont pas acceptables. Alors que les images et les vidéos pornographiques banalisent les violences sexistes et sexuelles, les établissements scolaires doivent combattre celles-ci et contribuer à l'apprentissage d'un comportement comportement et d'une sexualité se pratiquant dans le respect des autres et de soi. Les lieux d'enseignement sont des places privilégiées pour sensibiliser chacune et chacun aux violences faites aux femmes, aux violences sexistes et sexuelles. Ces violences se pratiquent dans les établissements scolaires et prennent de très nombreuses formes, comme le montre le dossier de « Sexisme à l'école, silence dans les rangs », qui dénonce des attouchements sexuels et d'autres formes de violence. Afin d'endiguer ces violences sexistes et sexuelles et les violences faites aux femmes, il est nécessaire que, dès le plus jeune âge et tout au long de leur scolarité, les élèves y soient sensibilisés. Sans cet enseignement, les violences sexistes et sexuelles se perpétueront. Il s'agit dès lors de prendre en compte cette problématique pour mieux éduquer nos enfants. L'école est le lieu idéal pour le faire, parents étant quelquefois complètement démunis. Nous ne pouvons pas combattre les actes dans les cours d'école, de collège ou de lycée, et plus largement dans la société, si nous ne formons pas les élèves.

Par ces séances d'information et de sensibilisation, nous éduquerons les élèves au respect d'autrui et nous leur apprendrons à détecter, combattre et empêcher la reproduction de ces violences. Grâce à cette sensibilisation, les jeunes seront alors plus à même de repérer les violences faites aux femmes, les violences sexistes et sexuelles et de prévenir les équipes pédagogiques ou toutes les personnes ressources qui sont présentes dans les établissements. De la même manière, les élèves seront pour repérer les violences en dehors des établissements scolaires et les combattre. C'est aussi un outil pour les professeurs, qui sont souvent démunis face à la violence des rapports entre les garçons et les filles, un phénomène qui les submerge.

de l'éducation à la sexualité, qui traite dès l'école primaire de la prévention des violences sexistes et sexuelles, en application notamment d'une circulaire du 12 septembre 2018.

présenté par Mme Jasmin. Ces thématiques sont également abordées dans le cadre de l'éducation à la sexualité et de l'éducation morale et civique.

permettra de renforcer l'effectivité de la formation obligatoire des personnels éducatifs à l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, de garantir le caractère transversal et intégré de l'enseignement de l'égalité des sexes et, enfin, de doter la grande cause du quinquennat de leviers supplémentaires d'action à l'intention des jeunes générations.

de faire acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité, autant de sujets qui me semblent pleinement inclure l'égalité entre les hommes et les femmes. En outre, ce même code, dans son article L. 121-1, charge les écoles, collèges et lycées de contribuer à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Cet amendement me semble donc déjà largement satisfait,

dans ses dispositions générales, l'égalité entre les femmes et les hommes comme une mission fondamentale de l'école. C'est le sens notamment des articles L. 121-1 et L. 312-17-1, qui disposent que l'école contribue, à tous les niveaux, à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation, ainsi qu'à prévenir les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. Cette exigence de transmission du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes se fait dès la formation dans les écoles élémentaires. Elle se fonde en particulier sur l'enseignement moral et civique, qui fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de la laïcité. que de la laïcité. Cela fait partie intégrante des missions des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, qui doivent « sensibiliser l'ensemble des personnels enseignants et d'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations ». Ces principes et cette ambition pour l'école trouvent une déclinaison concrète dans les objectifs et les mesures définis par la convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif, que nous allons renouveler pour la période 2019-2024, et qui constitue un important levier pour mettre en oeuvre auprès des jeunes générations la politique d'égalité entre les femmes et les hommes, définie comme la grande cause du quinquennat. Ce texte-cadre s'attache à développer une approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes, en articulant les enjeux de pilotage de formation, d'éducation, d'orientation et de lutte contre les violences.

La commission a considéré que la formation scolaire devait préparer l'élève à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme et de citoyen.

Le présent amendement vise à intégrer la dimension environnementale dans le partage des valeurs de la République comme mission première du service public de l'éducation. Les dispositions générales du code de l'éducation sont ainsi enrichies de la notion de respect et de préservation de l'environnement, au même titre que la dignité des êtres humains. Cet alignement de valeurs est indispensable pour préparer les jeunes générations aux profonds changements qui les attendent en matière de transition écologique. Il répond également à une attente légitime de leur part sur le rôle de l'institution éducative comme relais de diffusion des valeurs écologiques. Placer la préservation de l'environnement au même niveau de valeur que la dignité humaine est un symbole fort envoyé aux élèves et à leur famille. C'est aussi un outil supplémentaire, afin de renforcer la transmission de moyens concrets pour agir favorablement sur leurs environnements directs et de penser la transition écologique de manière globale. Quel est l'avis de la commission ?

des jeunes, notamment des lycéens, le 15 mars dernier. Comme vous le savez, nous avons organisé des débats dans les lycées à cette occasion, qui se sont poursuivis par d'autres débats, jusqu'à

j'ai invité mes collègues du Gouvernement chargés de l'environnement. Ce moment a été extrêmement fructueux et utile. Nous en tirerons toute une série de conséquences à la fois sur les contenus des programmes et des formations, mais aussi et surtout sur l'action quotidienne de nos élèves en matière d'environnement.

De proche en proche, nos 12 millions d'élèves peuvent considérablement contribuer à mener des luttes concrètes au service de l'environnement. Tout cela va évidemment dans le sens de votre proposition.

C'est pourquoi tout enfant a droit à une éducation manuelle, car c'est un levier puissant pour comprendre, apprendre, progresser et se construire. En effet, la main et le cerveau sont liés et travaillent ensemble. Nous sommes nés de cela,

De plus, comment un élève qui n'a pas la chance d'avoir des parents artisans ou bricoleurs, qui donc n'a pas vu, senti, vécu ni essayé le travail manuel, et qui n'a plus goût à l'école peut-il savoir qu'il est fait pour

alors certains que leur accomplissement est là. Au-delà, ce serait pour tous nos élèves l'occasion unique d'aller vers plus d'autonomie en réalisant un projet concret de A à Z. Fabriquer un objet, un vêtement, apporte satisfaction et fierté, mais aussi une forme d'humilité.

Sur le fond, je suis pleinement d'accord avec Angèle Préville : la formation scolaire ne fait pas une part suffisante à l'intelligence de la main.

revaloriser le travail manuel, non seulement pour les meilleurs, pour ceux qui excellent en lycée professionnel ou en apprentissage dans les métiers manuels, mais aussi pour l'ensemble des élèves, quelles que soient les orientations qu'ils prendront ensuite. C'est pourquoi dès l'école primaire et au collège

qu'il en soit, la référence au sein du code de l'éducation à l'éducation manuelle est saine et me paraît de bon aloi pour permettre des évolutions futures, afin de progresser concrètement en la matière. Aujourd'hui, et contrairement à d'autres sujets que nous avons abordés jusqu'à présent, cette référence est insuffisante. C'est pourquoi je suis favorable à votre proposition.

aussi à l'âge adulte. Or ces activités apportent épanouissement et sérénité. C'est donc un bien pour la société tout entière, une richesse qui, avec le sport et la culture, constitue un viatique vers une certaine forme de bonheur. Kant disait car c'est dans le problème de l'éducation que gît le grand secret de la perfection de la nature humaine » ! La parole

il s'est fait massacrer par le système scolaire. Il est arrivé à la ferme totalement dévalorisé, exerçant une profession qu'on lui avait mise dans les mains et qui ne lui plaisait pas. Il n'a pas véritablement choisi son orientation. Mon associé et

plus d'égalité dans notre République en favorisant également l'éducation manuelle ? La parole